à la charge du professionnel condamné les frais relatifs à l’assistance à laquelle l’association de défense des consommateurs peut recourir pour le traitement des demandes d’indemnisation des membres du groupe. Il s’agit de généraliser cette faculté à toutes les actions de groupe et de faciliter la mise en œuvre de ces procédures en réduisant le coût pour le demandeur de la phase de liquidation des préjudices.

et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur, n’est en effet qu’un leurre. Certes, l’entreprise mise en cause ne pourrait plus disposer de cet argent destiné à indemniser les victimes, mais ces dernières ne toucheraient pas non plus l’indemnisation. Compte tenu de la longueur des procédures d’action de groupe, voilà qui est inacceptable. C’est pourquoi nous demandons que le jugement sur la responsabilité soit exécutoire à titre provisoire, comme le prévoit le code de procédure civile. Quel

revenir au droit en vigueur, en prévoyant que les mesures de publicité ne sont applicables qu’à l’extinction des éventuels recours ordinaires et pourvoi en cassation. En outre, il paraît dommageable de retirer au juge la possibilité d’ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur,

effet, comme vous l’avez d’ailleurs très bien rappelé, le droit commun dispose d’ores et déjà que les décisions de première instance sont par principe exécutoires. Ces dispositions s’appliqueront naturellement au jugement statuant sur la responsabilité du défendeur dans le cadre d’une action de groupe. Par ailleurs, il nous semble important de conserver les dispositions de l’article 1 tel qu’il est rédigé actuellement

du code monétaire et financier est particulièrement clair : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. » Je ne suis donc pas favorable à ce que de telles sommes soient conservées par des notaires ou des avocats. La commission demande le retrait de cet

qu’, en cas d’accord. Dans le cas spécifique des actions de groupe, la médiation est marquée, elle aussi, par le déséquilibre entre la partie demanderesse et la partie défenderesse. La première est généralement une association, dotée de moyens très limités, qui, de surcroît, ne dispose pas de toutes les informations sur le litige. La seconde est fréquemment une entreprise qui dispose de davantage de ressources

Plus spécifiquement, nous souhaitons éviter que la partie défenderesse ne profite de la médiation pour mettre certains frais à la charge de l’autre partie. En effet, la loi dispose actuellement que la répartition des frais est librement déterminée par les parties. Compte tenu du déséquilibre que j’ai évoqué, qui est souvent considérable, on pourrait imaginer une situation dans laquelle une entreprise conditionnerait l’accord de médiation à la prise en charge d’une partie des frais afférents par l’association demanderesse. Certes, le juge pourrait s’opposer à une telle répartition des frais lors de la vérification de l’accord, mais il ne serait pas tenu de le faire. Ainsi existe t il un risque financier potentiellement important ; en particulier, de petites associations, de réserves financières très limitées, pourraient se trouver dissuadées d’introduire des actions de groupe. Or notre objectif est de faciliter les actions de groupe. Vous l’aurez deviné, mes chers collègues : le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite, par le biais de cet amendement, interdire que les frais de la médiation soient mis à la charge de la partie demanderesse.

Le droit commun de la médiation, applicable aux procédures de médiation engagées dans le cadre d’une action de groupe, prévoit, certes, que les parties déterminent librement la répartition des frais de médiation. En l’absence d’accord entre les parties, les frais sont théoriquement répartis à parts égales. Le juge peut néanmoins estimer que cette répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties et, en conséquence, décider d’une autre répartition. Il existe donc déjà des mécanismes, à la main du juge, permettant de protéger les associations, dont les budgets sont plus contraints que ceux des entreprises. En deuxième lieu,

à ce que les frais occasionnés par une action de groupe en réparation soient mis à la charge de la partie perdante. Il ne traite donc pas des frais de médiation. En troisième lieu, une médiation est une procédure amiable

procédure et qu’il est « envisageable d’imposer au juge de mieux prendre en compte, au titre de l’appréciation des frais non compris dans les dépens la réalité du travail fourni par l’association et son conseil juridique qui peut varier sensiblement en fonction de la difficulté de la preuve de la responsabilité de l’entreprise et de la taille du groupe des victimes ». En résumé, la justice a un coût et la réussite des actions de groupe ne fait pas exception.

de se faire connaître pour se rallier à la plainte, devraient être à la charge du défendeur. Cette mesure est rendue légitime par le fait que le juge a déjà admis à ce stade la responsabilité du défendeur. Notre proposition est d’autant plus importante que les subventions de l’État aux associations de consommateurs ont connu une forte baisse ces dernières années, passant de 3,64 millions d’euros en 2014 à 2,83 millions d’euros en 2019. Par exemple, la subvention à la Confédération nationale du logement est passée de 219 952 euros en 2014 à 185 512 euros en 2018. l’UFC Que Choisir a perdu plus de 100 000 euros sur la même période. Nous pensons qu’il faut inverser la responsabilité financière.

devant l’ensemble des juridictions sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le retentissement médiatique d’une action engagée peut avoir des effets considérables, voire destructeurs,

avant le prononcé du jugement ou lorsque l’action de groupe a fait l’objet d’un désistement, irait à l’encontre de la présomption d’innocence. La publicité donnée en effet d’être assimilée à un prononcé sur la responsabilité du professionnel. Pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas les moyens de se défendre, il est proposé que les actions

Le registre mis à la disposition du public, qui est tenu par le garde des sceaux, recense les actions de groupe, les actions en reconnaissance de droit et les actions collectives. Je suis opposé à la suppression pour plusieurs raisons. D’abord, l’objectif principal de la création de ce registre est précisément d’améliorer l’information des justiciables pour leur permettre, part, de rejoindre plus facilement ces actions lorsqu’ils sont concernés et ainsi de favoriser l’indemnisation des victimes ; d’autre part, de savoir quelles actions ont prospéré dans le passé pour estimer si leur propre initiative est elle même susceptible de prospérer. Supprimer la publicité de ce registre le rendrait en fait inutile. Ensuite, la commission a précisément souhaité étendre le contenu de ce registre pour parfaire l’information des justiciables. La suppression de la mise à disposition de ce registre est donc contraire à la position de la commission, raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre

J’ai encore entendu hier, à Aix en Provence, le garde des sceaux décliner cet objectif, que nous partageons. D’ailleurs, le Gouvernement a annoncé récemment que les convocations au tribunal ne devront plus obliger la personne convoquée à se rendre disponible pendant toute

La deuxième, c’est qu’au regard des spécificités de la procédure et des domaines juridiques concernés, seule une spécialisation poussée des magistrats et des greffiers sur quelques tribunaux permettra de donner du sens à cette spécialisation.

opérant en matière d’action de groupe dans la mesure où, d’une part, l’action de groupe est portée par un seul demandeur – une association au nom de l’ensemble des membres du groupe – et, d’autre part, elle concerne potentiellement des justiciables répartis sur l’ensemble du territoire national,

l’augmentation des budgets, le stock des affaires en traitement, qui se sont accumulées, reste très important. En matière civile, par exemple, il faudrait 637 jours à nos juridictions pour traiter toutes les affaires pendantes, alors qu’il en faudrait seulement 237 selon la médiane européenne. Dans ce contexte, tout gain d’efficacité devrait être bon à prendre. C’est ce que le groupe écologiste propose par le biais de cet amendement qui vise à ce que la juridiction qui statue sur une action de groupe en matière environnementale puisse également statuer sur la réparation du dommage écologique. Même si cela pourrait paraître logique, ce n’est pas ce que le texte prévoit en l’état. En effet, outre la cessation du manquement, l’action de groupe ne peut viser que la réparation du dommage subi par les personnes lésées composant le groupe.

partage en tout point l’avis de la commission. Tout d’abord, l’action de groupe prévoit que la réparation est directe et intégrale pour les seuls préjudices subis par les personnes membres du groupe.

En effet, les avocats jouissent d’un monopole s’agissant de l’assistance et de la représentation des justiciables devant les juridictions. Pour les autres activités d’accompagnement juridique, hors des tribunaux, les justiciables sont libres de choisir le professionnel du droit de leur choix : un avocat, un notaire ou un commissaire de justice. Il n’apparaît donc pas nécessaire de rappeler dans la loi une faculté offerte aux demandeurs d’une action de groupe. L’amendement

Tout d’abord, indépendamment de toute disposition législative, le demandeur, s’il le souhaite, pourrait s’adjoindre les services d’un avocat pour l’assister dans la phase de liquidation des préjudices. En outre, d’autres professions judiciaires réglementées, comme les commissaires de justice, répondent aux exigences d’expertise et de déontologie, leur permettant d’exercer cette mission particulière d’assistance auprès des associations. Ainsi, le Gouvernement serait favorable à la réintroduction de l’article 2 A sous réserve de deux aménagements : l’élargissement à d’autres professions judiciaires réglementées, comme les commissaires de justice

qui peut introduire une action de groupe ? Cette question est essentielle, mais la problématique de la qualité pour agir ne se pose pas seulement au moment de l’introduction d’une action de groupe. En effet, la qualité pour agir pourrait se perdre, pour une raison ou une autre, au cours de la procédure. On pense ici, bien évidemment, à l’association Anticor, qui a perdu en décembre dernier l’agrément qui lui permettait de se constituer partie civile. Nous risquons de rencontrer des situations similaires pour les actions de groupe. Or, dans l’intérêt des personnes lésées, il est primordial que les procédures entamées puissent être menées à leur terme. personnes ont potentiellement déjà investi du temps pour suivre l’action de groupe et espèrent pouvoir toucher une indemnisation pour le préjudice subi. Leur annoncer que l’action de groupe se termine du jour au lendemain risquerait d’éroder la confiance dans cette procédure. De plus, il faut rappeler que la perte de la qualité pour agir ne dit rien sur la responsabilité de la personne mise en cause. De même, elle ne dit rien sur les modalités d’une indemnisation dans le cas où la responsabilité serait reconnue. Ces questions seront appréciées par les tribunaux. Les magistrats spécialisés, qui statueront sur les questions pendantes, Les magistrats spécialisés, qui statueront sur les questions pendantes, méritent notre pleine confiance. Enfin, notre proposition entend limiter les conséquences d’une décision politique, alors que les actions de groupe devraient rester en dehors de toute ingérence de ce type. Nous voulons simplement garantir que les actions en cours soient menées à leur terme.

déjà satisfait par la rédaction actuelle de l’article 2, lequel dispose qu’en cas de défaillance du demandeur « toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur ». Dans ces conditions,

Comme nous l’avons souligné lors des débats sur les médiations, cette charge financière peut amener associations et syndicats à renoncer à introduire une action de groupe. Ce risque financier, quelque peu absurde, s’explique par le fait que le code de procédure civile serait applicable aux actions de groupe en matière civile. Sur le

De plus, la Cour de cassation a également établi le principe que la condamnation au paiement des frais de procédure n’est pas conditionnée à la reconnaissance d’une faute. Il existe donc un réel risque, dans certains cas, l’action de groupe soit considérée comme relevant d’une « procédure trop lourde » et que l’association ou le syndicat soient amenés à régler une partie des frais de procédure. Cela irait à l’encontre de l’esprit de la directive européenne de 2020 sur les actions de groupe, qui demande aux États membres de veiller à ce que des considérations financières

dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

S’enrichir en transgressant la loi, voilà une situation que nous voulons toutes et tous ici éviter. Pour autant, elle peut se produire si les sanctions des infractions sont moins élevées que les gains économiques que leurs auteurs peuvent en tirer. Ce risque est particulièrement élevé pour les fautes qui donnent lieu à une action de groupe, laquelle permet uniquement de réparer le préjudice subi.

le montant de la condamnation [soit] très probablement inférieur au profit retiré par l’entreprise du fait du non respect des dispositions légales ou contractuelles ». Dans de telles situations, l’entreprise serait encouragée à transgresser la loi, à mettre son devoir de vigilance de côté.

anormal qu’un professionnel puisse volontairement commettre des manquements dans le seul but d’en tirer des gains illicites, sans craindre des pénalités financières. Le législateur, de même que le pouvoir judiciaire, est là pour moraliser la

Il est défendu. à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, au lieu de 5 %. Cette mesure, proposée par les députés ayant rédigé le rapport d’information et la présente proposition de loi, est également préconisée par la Défenseure des droits dans son avis sur le texte. On pourrait même réfléchir à flécher le produit de cette sanction vers les associations habilitées à introduire une action de groupe.

Premièrement, la proposition de loi que nous avons à examiner ce soir vise à unifier le régime des actions de groupe et à transposer la directive européenne du 25 novembre 2020. Or la sanction civile n’est pas imposée par le droit européen. Deuxièmement, la création d’une sanction civile constitue une réforme d’ampleur du droit de la responsabilité civile, qui mériterait d’être discutée, à mon sens, dans un autre cadre. Troisièmement, la sanction civile ne fait pas consensus entre les tenants de la doctrine, les praticiens du droit et les acteurs économiques. Ces derniers y sont – pour la plupart – particulièrement opposés, comme l’ont rappelé les personnalités que j’ai pu auditionner. En outre, lorsque la commission des lois a étudié cette sanction civile, elle s’est toujours montrée très réservée sur sa création dans notre droit interne. Quatrièmement, tant le Conseil d’État que la direction des affaires civiles et du sceau ont fait part de leurs réserves, voire de leur opposition à la création d’une amende civile, à la fois pour des raisons de forme – je viens de les évoquer – et de fond.

le principe d’un cumul possible de cette sanction avec une amende administrative ou pénale, mais la rédaction retenue est trop générale et ne donne pas les leviers nécessaires au juge pour apprécier de manière précise la proportionnalité d’une telle sanction.

doivent être mises à disposition du public dans toutes les langues de l’Union européenne pour pouvoir exercer des actions de groupe transfrontières. Une telle précision ajouterait une nouvelle obligation non prévue par la directive et ne serait donc pas conforme au droit européen.

En effet, c’est la Commission qui veille à ce qu’aucune situation potentiellement problématique ne se produise. À ce titre, elle peut, par exemple, demander à l’Autorité de la concurrence et à ses homologues des autres pays membres de vérifier si les associations qui peuvent entamer une action de groupe transfrontalière ne violent pas les conditions pour le faire.

Pour cette raison, la directive européenne demande explicitement que la Commission européenne soit informée de toute modification du registre des acteurs habilités. En toute logique, les États membres ayant déjà transposé cette directive ont également inscrit dans leur droit cette obligation d’information, à l’instar du Portugal.

pourraient toujours être engagées en matière de lutte contre les discriminations sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, mais elles seraient soumises au régime procédural antérieur. Les

D’une part, parce que nous sommes déjà en retard : la France, comme tous les États membres de l’Union européenne, avait jusqu’au 26 décembre 2022 pour transposer la directive européenne sur les actions de groupe.

pour les actions de groupe en matière de discriminations ou de questions environnementales, sans que le Conseil constitutionnel ait à s’en émouvoir particulièrement. D’autre part, il existe déjà des différences entre le justiciable recherchant la réparation du préjudice à titre individuel et celui la recherchant à titre collectif,

Ensuite, à supposer qu’un opérateur n’étant pas en situation de manquement n’ait pas à craindre une action de groupe, il n’en demeure pas moins que les contrats d’assurance le couvrant en cas de réalisation de ce risque – qui ne résulte pas toujours d’une intention malveillante – ne

pas le fond du droit de la responsabilité n’enlève en aucun cas le coût réputationnel important que peut induire sur un opérateur, y compris de petite taille, une action de groupe.

Or, pour revenir à la problématique de l’assurance, les contrats de protection juridique de ces personnes n’ont logiquement pas été calibrés à cette fin, dans des domaines qui n’y étaient jusqu’à présent pas soumis. Le coût qui va en résulter ne saurait être mésestimé.